Plusieurs de mes collègues étaient et sont toujours hostiles au passe, tout en étant très ouvertement favorables à la vaccination, mais une large majorité des sénateurs centristes a voté en faveur de son déploiement en juillet dernier.

Madame la ministre, les rapports, c'est bien, mais le vote de la représentation nationale nous semble préférable ! Le Parlement, et le Sénat en particulier, a toujours répondu présent depuis le début de la crise sanitaire, y compris lorsqu'il a dû délibérer dans l'urgence absolue. Nous entendons continuer à exercer exercer pleinement notre rôle de législateur et notre mission de contrôle de l'action du Gouvernement. Le Sénat refusera, je le répète, de jouer à la roulette russe avec des mesures d'urgence.

en réduisant significativement les risques de contamination et les cas graves. La pression hospitalière se fait plus faible. C'est pourquoi je comprends que l'on puisse s'interroger sur l'utilité des dispositifs liés à la gestion de cette crise. En disant cela, je ne nie pas le risque de rebond épidémique qui, je le sais, persiste malgré la vaccination. Mais je m'interroge sur l'intérêt qu'il y a à voter la prorogation d'un régime exceptionnel, de manière systématique, et pour des durées toujours plus longues.

Il l'est d'autant plus qu'en avril dernier le Président de la République déclarait que ce passe sanitaire ne serait jamais un droit d'accès qui différencie les Français, et qu'il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas.

viendra apaiser certaines incompréhensions. Si certains membres de notre groupe restent fondamentalement opposés au passe sanitaire, ces aménagements sont de nature à en rassurer d'autres. Enfin,

Il faut espérer qu'un consensus se dégage à ce sujet. Nos institutions doivent en effet pouvoir s'entendre sur des enjeux aussi importants et ne pas montrer leurs divisions et leur dispersion, notamment à quelques mois d'une période électorale majeure, pendant laquelle les populismes les plus nauséabonds devront être combattus.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après vingt mois d'impréparation, d'erreurs et de mensonges, j'ai découvert cette nuit que le Gouvernement avait radicalement changé d'orientation. Après l'annonce tant attendue de la démission du ministre de la santé, le Parlement décide enfin d'en finir avec le passe sanitaire le 15 novembre prochain et fait sauter l'obligation vaccinale, tout comme celle du port du masque. L'état d'urgence permanent qui nous est imposé depuis dix-huit mois, avec une affligeante docilité parlementaire, est enfin abandonné. Pour lutter contre la résilience de la maladie, le traitement et la prise en charge du covid long sont actés. La recherche d'un traitement est privilégiée, en même temps que le soutien aux vaccins français. La chaîne industrielle nationale et indépendante, qui doit nous garantir un approvisionnement sans pénurie, est désormais une priorité. Les moyens humains nécessaires aux contrôles aux frontières sont débloqués pour mieux contenir les résurgences épidémiques. Après des années de saccage de l'hôpital public, un grand plan pour nos hôpitaux et nos personnels soignants sera présenté par le nouveau ministre de la santé dans la journée. L'application TousAntiCovid, coûteuse et dangereuse, et les contrôles numériques sont proscrits, les verbalisations et les tests payants abandonnés. Le chef du Gouvernement annonce même, je le cite : « Nous avons écouté, nous avons entendu le peuple français. Ainsi, la loi redevient légitime : orientée vers l'unité du peuple et le bien commun ». Les visages, les sourires, le contact, la simplicité, la confiance, l'esprit de voisinage et de communauté sont de retour. La France est de retour Je n'ai pu, mes chers collègues, retenir un large sourire de satisfaction, en même temps que coulaient sur mes joues des larmes d'émotion. Oh ! Oh ! Et puis ... mon réveil a sonné et je me suis réveillé De ce retour à la liberté il n'est nullement question : le Parlement est toujours aussi docile et l'sanitaire sera, j'en ai bien peur, reconduit. Le chantage à la vaccination est confirmé

Le seul qui soit sur la sellette, ce n'est pas le ministre de la santé qui se sera trompé ou qui aura menti depuis le début de la crise sanitaire. Non ! Raoult ! Le seul sur qui les pouvoirs publics et pharmaceutiques s'acharnent aujourd'hui, ... Raoult ! ... c'est le professeur Raoult ! Cet irréductible gaulois Cet irréductible gaulois de la médecine, qui aura commis le seul crime de soigner à un coût dérisoire, est aujourd'hui lâché par des élus dont je tairai le nom, qui, alors qu'ils étaient atteints du covid, se sont précipités à l'institut hospitalo-universitaire de Marseille pour bénéficier du traitement de celui qu'ils traînent aujourd'hui dans la boue. En les écoutant, on ressent le besoin urgent d'un traitement contre la nausée Ces libertés retrouvées n'étaient donc qu'un rêve, le songe d'une nuit d'automne. Il ne tient pourtant qu'à nous, mes chers collègues, d'en faire une réalité. Tel est l'espoir de la France et des Français ! Puissiez-vous enfin les écouter

Monsieur le président, madame la ministre,

Pour la onzième fois en vingt mois, nous nous apprêtons à examiner un texte visant à faire face à la crise sanitaire. Et pour la onzième fois, l'exécutif nous pousse à examiner à la hâte un texte qui, pourtant, touche au coeur de nos libertés publiques et de nos droits les plus fondamentaux. Ce qui pouvait, au début de la pandémie, se justifier par l'urgence peine aujourd'hui à s'expliquer, soit par un manque d'anticipation, soit par une absence de considération du rôle du Parlement- j'y ai fait référence en préambule Que propose le Gouvernement ? Rien de moins que de prolonger jusqu'à l'été 2022, c'est-à-dire au-delà de la fin du quinquennat, le cadre juridique permettant de déclarer l'urgence sanitaire ou le régime transitoire aujourd'hui Parce qu'il dessaisit le Parlement pour une durée au-delà de l'acceptable, par ce qu'il impose pour une durée exceptionnelle et excessive au regard de la nécessité, ce projet de loi porte atteinte au bon fonctionnement de notre démocratie. Pourquoi faudrait-il proroger l'état d'urgence pour si longtemps ? La tenue d'élections, aussi essentielles pour notre démocratie soient-elles, ne peut pas être un motif valable. Rappelons que le Parlement peut toujours être réuni, à tout moment si besoin. Quand bien même nous ne partagions pas les orientations du Gouvernement, nous avons toujours fait preuve de réactivité et su nous mobiliser ; nous avons largement prouvé notre capacité à voter un tel régime dans une temporalité très courte. En mars 2020, vous vous en souvenez, nous l'avons fait dans des conditions que l'on pourrait qualifier d'extrêmes, en plein confinement. La situation sanitaire n'est aujourd'hui plus la même : le taux d'incidence est désormais inférieur au premier seuil d'alerte dans presque tous les départements, et la covid-19 fait partie de notre quotidien. Je reprends d'ailleurs l'argument très juste de mon collègue Bernard Jomier. Lors de l'audition du ministre de la santé,

Aussi, si nous devons apprendre à vivre durablement avec le virus, nous devons le faire dans un régime de droit commun. Nous ne pouvons accepter de prolonger aussi durablement un régime d'exception, qui porte profondément atteinte à l'État de droit. Nous ne devons pas nous habituer à vivre dans une société où les libertés Il apparaît au contraire nécessaire de nous interroger régulièrement, au vu de la situation, pour savoir si ces restrictions sont toujours justifiées. Ces questionnements n'ont pas manqué de traverser les rangs mêmes de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Je pense évidemment à l'amendement du député Marche Pacôme Rupin, adopté en commission, qui tend à circonscrire l'utilisation du passe sanitaire aux départements dont le taux d'incidence du virus dépasse les 50 cas pour 100 000 habitants par semaine. Mais au-delà, soulignons que ce projet de loi n'a été adopté que d'une très courte majorité- 10 voix -à l'Assemblée nationale.

Le passe sanitaire ne représente plus aujourd'hui un levier efficace pour convaincre le reste de la population éligible de se faire vacciner. Se pose dès lors la question légitime de la prolongation d'un dispositif, qui a épuisé tous ses effets d'incitation à la vaccination,

Notre objectif est toujours le même : celui d'une vaccination universelle, solution que le Gouvernement et la majorité sénatoriale ont rejeté en juillet et en octobre, et qui est pourtant la seule solution claire, durable et transparente. Il est dès lors de la responsabilité du Gouvernement de trouver les moyens de convaincre les plus réticents de se faire vacciner et de conduire une éventuelle campagne de rappel, campagne qui semble même avoir commencé pour une partie de la population, bien que certains arbitrages se fassent toujours attendre. Le passe sanitaire intégrera-t-il cette troisième dose de rappel ? Sera-t-elle obligatoire pour les soignants ? À ce jour, le ministre de la santé n'est pas capable de répondre Sur ces différents sujets, le Gouvernement peine à fournir des éléments précis et à rétablir un climat de confiance, tant avec la représentation nationale qu'avec les Français. Notre groupe s'oppose également à la disposition introduite par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, qui autorise les chefs d'établissement du primaire et du secondaire à

Mes chers collègues, encore une fois, la méthode n'est pas à la hauteur du débat que méritent les Français. Le contenu du texte suscite bien plus d'inquiétudes qu'il n'en calme, alors même que la situation sanitaire nous laisse entrevoir un retour prochain à une vie normale. Nous vivons avec cette pandémie depuis maintenant de nombreux mois. Même si tout le monde en est un peu lassé, le port du masque, les gestes barrières et les mesures visant à freiner la propagation de l'épidémie sont toujours largement acceptés et suivis. Dans le même temps, la couverture vaccinale a beaucoup progressé. La lutte contre la pandémie va dorénavant s'inscrire dans un temps extrêmement long. Le moment est largement venu de retrouver nos libertés fondamentales et de renouer avec l'État de droit. C'est un enjeu pour notre démocratie et pour la République. La position du groupe socialiste est claire nous refusons d'accorder un blanc-seing pour une période qui enjambe deux élections nationales majeures. Toute restriction des libertés doit relever de la seule compétence du Parlement. Oui ! En cela, nous partageons l'analyse du rapporteur, qui vient encore de le manifester de manière expressive. Nous refusons également que les directeurs d'école puissent connaître le statut vaccinal de leurs élèves. Oui ! Nous refusons la prolongation de toute forme de passe sanitaire dans les territoires où il n'est plus nécessaire.

M. le rapporteur, nous nous sommes retrouvés onze fois depuis le début de cette pandémie. Jamais un parlement en Europe n'a été autant sollicité ! C'est bien la démonstration que le Gouvernement est toujours à l'écoute de nos deux chambres. le rapporteur, notre compréhension, notre analyse et les outils en notre possession ont considérablement évolué depuis mars 2020. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui avec des mesures bien moins restrictives que le couvre-feu ou le confinement. Nul ne niera, par exemple, que le passe sanitaire a fait ses preuves. Déposé le 13 octobre 2021, le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire vise à proroger le régime de sortie de crise sanitaire, donnant au Gouvernement la faculté de mobiliser une gamme d'outils de gestion de la crise si la situation l'exigeait, y compris de manière territorialisée, et ce, sous le contrôle du juge et sous le contrôle, renforcé lors de l'examen à l'Assemblée nationale, du Parlement. mesures importantes : le report au 31 juillet 2022 de la fin du cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire, fixée aujourd'hui au 31 décembre 2021

la facilitation du contrôle de l'obligation vaccinale et le renforcement de son efficacité ; enfin, la prorogation de plusieurs mesures d'accompagnement pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, le dispositif d'activité partielle

Cette situation, il faut en parler. Après huit semaines de baisse consécutive, le taux d'incidence a augmenté de 10 % durant la semaine du 10 au 17 octobre. Conséquence, le pays a dépassé le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a, quant à lui, franchi la barre symbolique des 5 000 cas depuis trois jours. À l'approche de l'hiver, les épidémiologistes gardent tous les yeux rivés sur les courbes. Nous devons collectivement faire de même. Pour autant, 7 millions de Français ne sont pas encore convaincus. Si, en France, « les voyants virent au orange », comme le titrait hier, la carte de l'Europe, quant à elle, se colore de rouge. Le nombre de cas de covid-19 recensés chaque jour a augmenté d'une semaine à l'autre dans la quasi-totalité des pays du continent. La tendance est générale des cas en Italie, de 48,5 % en Allemagne, de 57 % en Autriche, avec des pointes à 95 % en Pologne, et même à plus de 120 % en République tchèque. À cela s'ajoutent la contagiosité accrue du variant delta, le ralentissement de la progression de la couverture vaccinale et la baisse progressive de l'efficacité de la protection du vaccin au fil du temps, en particulier chez les personnes âgées, premières cibles de la campagne. enfin la possibilité de l'émergence de nouveaux variants, avec des facteurs de risque plus importants ou une moindre sensibilité aux vaccins disponibles. À cet égard, le Royaume-Uni et son nouveau sous-variant nous invitent à la vigilance.

Or, en application du texte de la commission, non seulement les mesures de freinage seraient agencées dans une nouvelle architecture bien complexe, mais le passe sanitaire ne pourrait plus être mis en oeuvre dans les départements où le taux de vaccination de la Faut-il rappeler que plus de 75 % de la population du Royaume-Uni est vaccinée ? Voilà pour les chiffres. Mais il n'y a pas que les chiffres. Pensons aux personnels soignants, épuisés par le travail extraordinaire qu'ils ont réalisé depuis deux ans. Ils veulent de la stabilité et de la clarté dans les mesures proposées. Changer notre fusil d'épaule juste avant la saison hivernale ou dans quatre mois ne leur rendrait pas service. Ce texte doit nous permettre d'accélérer encore la vaccination. Regardons au-delà de nos frontières : en Allemagne, certains autorisent désormais les restaurateurs et les exploitants de lieux culturels à refuser les non-vaccinés, bien que testés négatifs ; en Autriche, si la situation s'aggrave, seuls les habitants non vaccinés pourraient faire l'objet d'un confinement. Que dire de la Chine, qui reconfine 4 millions de ses habitants ? Personne, en France, ne souhaite en arriver là. Il s'agit non pas d'accoutumance, mais de prévention. Il s'agit non pas de donner un blanc-seing au Gouvernement, mais de lui conférer l'agilité nécessaire pour faire face à une pandémie qui a mis le monde entier à genoux. Il s'agit de s'adapter à la rapidité avec laquelle le virus continue de nous surprendre, au même titre que la Chambre Haute a su s'adapter à plusieurs reprises,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suppose que vos boîtes mail ont été une fois de plus envahies, comme la mienne, par les milliers de spams envoyés par les antivax, les antipasse et, plus généralement, les « anti-tout-ce-qui-bouge » ! Robert Kennedy avait coutume de dire : « un cinquième des gens sont contre tout, tout le temps Je voudrais commencer par dire à ces trolls que les campagnes de spams déclenchent chez moi une réaction quasi-réflexe : l'envie de voter dans le sens opposé à ce qu'ils demandent, ou plutôt exigent. Je ne pense pas être le seul La quatrième vague, due au variant delta, qui est trois fois plus contagieux que la souche initiale, régresse depuis deux mois grâce à trois mesures : la vaccination massive, le respect des gestes barrières et le passe sanitaire. La France est aujourd'hui l'un des pays, voire le pays au monde dont la population est la plus vaccinée, et cela lui permet d'être dans une situation très enviable, même si elle reste fragile. Nous savons désormais que le vaccin réduit de 92 % le risque d'hospitalisation chez les plus de cinquante ans. Ce chiffre finit de déconsidérer ceux qui, depuis des mois, tentent de discréditer la vaccination. dernière a fait ses preuves, le passe sanitaire aussi. Nous allons donc débattre des modalités de prolongation du passe sanitaire, et non du dispositif lui-même. Le passe est autorisé jusqu'au 15 novembre, c'est-à-dire dans quinze jours, et la grande majorité de cette assemblée n'a aucunement l'intention, pour l'heure, L'épidémie n'est pas finie : elle flambe à nouveau chez nos voisins et tous les scientifiques s'attendent à une recrudescence hivernale. Ne pas prolonger le passe serait une erreur majeure, n'en déplaise à ceux qui défilent au nom des libertés bafouées. La plupart des Français le comprennent et l'acceptent. Ils savent que les quelques désagréments liés au passe sont peu de chose par rapport à un reconfinement, si la situation devait s'aggraver. Ils ont bien saisi que le passe est un outil, non de contrainte, mais de liberté.

Le conseil scientifique l'approuve aussi et comprend la nécessité opérationnelle de cette durée, compte tenu de la persistance de risques potentiels jusqu'au 31 juillet. Ces arguments ont du poids, mais nous sommes des parlementaires, jaloux à juste titre de nos prérogatives et toujours rétifs, lorsqu'il s'agit des libertés, à nous en dessaisir pour de longues périodes. J'étais donc partagé sur ce sujet. Je ne le suis plus depuis que j'ai pris connaissance du texte de la commission, qui ne me paraît pas satisfaisant. D'abord, il est devenu illisible, et je ne suis pas le premier à le

à un mois de l'élection présidentielle, nous discuterons probablement de tout sauf des mesures contre l'épidémie. Enfin, nous avons besoin d'une réponse rapide en cas de nouvelle flambée. En juin dernier, c'est l'intervention immédiate du Président de la République, faisant le choix du passe sanitaire devant l'explosion de l'épidémie, qui a permis l'adhésion de tous les Français à la vaccination.

Chez la plupart de nos voisins, les mesures de lutte contre l'épidémie ont été prises par simple décret. En France, comme Philippe Bas l'a rappelé, c'est la onzième fois que le Gouvernement vient demander son autorisation au Parlement. Permettez-moi de penser, dans ces conditions, que les mines offusquées de ceux qui accusent l'exécutif de

nous achevons nos travaux de la semaine par l'examen d'un texte important, sur un sujet qui nous est désormais très familier : la gestion de la crise sanitaire. Le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire est d'ailleurs le onzième texte consacré à cette question, le Parlement ayant été amené, comme il se doit, comme il se doit, à se prononcer régulièrement sur le maintien, le renforcement ou l'assouplissement des différents dispositifs de lutte contre le virus. Chaque fois, le Sénat l'a fait dans une démarche de responsabilité à l'égard de nos concitoyens. Mais il l'a également fait en mesurant l'ampleur des perturbations que cela engendre dans la vie de nombre d'entre eux, en particulier les restrictions à certaines libertés que cela provoque. Pour ces raisons, notre assemblée a toujours été force de proposition et s'est efforcée, quand c'était possible, de parvenir à un compromis plus respectueux des droits et libertés des Français. Aujourd'hui, le Gouvernement revient vers nous avec un nouveau projet de loi. Son objectif est, pour l'essentiel, de prolonger l'application de la plupart des dispositifs actuels : le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le système d'information national de dépistage, certaines mesures administratives et économiques d'accompagnement, mais aussi et surtout, le passe sanitaire. Ce dernier fait débat tant parmi nos concitoyens qu'au sein de la représentation nationale. Sa mise en place, qui s'apparente à une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom, aura sans doute permis d'éviter un confinement supplémentaire, de faciliter la reprise d'un certain nombre d'activités et d'accélérer la vaccination, dont le taux atteint à présent un niveau élevé en métropole, ce dont nous pouvons nous féliciter.

À un moment où le taux de vaccination en France atteint un niveau élevé- 86 % des Français âgés de plus de 12 ans sont vaccinés -et où l'épidémie n'a plus l'intensité qu'elle pouvait avoir au début de l'été, il est légitime de songer à la sortie du passe sanitaire. Certains parmi nous ont plaidé en faveur d'une fin plus ou moins immédiate de son application. Ne pas souhaiter demeurer plus longtemps que nécessaire sous l'empire de ces dispositifs est compréhensible. Pour autant, la situation épidémique demeure fluide, et est susceptible de connaître des évolutions soudaines. Nous l'avons malheureusement constaté, le mois dernier, en Nouvelle-Calédonie. Le maintien d'un cadre robuste pour lutter contre la crise sanitaire est donc nécessaire. Le taux de vaccination, s'il est élevé sur le plan national, n'est toutefois pas homogène et reste comparativement faible par endroits. C'est le cas en outre-mer, dont les territoires ont été tout particulièrement éprouvés par l'épidémie durant les derniers mois. Pas plus tard que le mois dernier, nous votions le prolongement de l'état d'urgence sanitaire dans un certain nombre de territoires ultramarins. Aujourd'hui encore, le Gouvernement nous demande de maintenir l'état d'urgence sanitaire en Guyane et Martinique. La démarche de la commission des lois du Sénat a consisté à concilier ces différentes exigences : d'une part, ouvrir la voie à une sortie du passe sanitaire là où son application ne serait plus proportionnée

Ainsi, l'exécutif bénéficiera de prérogatives adaptées à la situation sanitaire actuelle. Il pourra maintenir le passe sanitaire dans une version atténuée, mais uniquement dans les départements où moins de 75 % de la population est vaccinée et où le virus circule activement. Par contraste, là où la situation s'est améliorée, le passe sanitaire ne s'appliquera plus. De cette manière, il sera possible de contrôler la propagation de la maladie là où il est nécessaire de le faire, tout en assouplissant les contraintes pesant sur les Français là où ces dernières ne seraient plus adaptées. Par ailleurs, en cas de dégradation de la situation, le Gouvernement pourrait, par décret et pour une durée limitée à un mois, disposer de prérogatives renforcées, inspirées pour partie du dispositif de l'état d'urgence sanitaire.

Pouvons-nous accepter que le Parlement ne se prononce plus sur ces problématiques relatives à la sécurité sanitaire et aux libertés fondamentales pendant plus de sept mois ? Pouvons-nous accepter d'enjamber ainsi des échéances électorales majeures dont le résultat est incertain ? Quel sera l'exécutif ? Quelle sera la majorité à l'Assemblée nationale ? Il ne serait pas responsable de prendre ce genre de risque. C'est pourquoi notre commission a décidé de ramener cette durée à trois mois et demi, en parfaite cohérence, une fois encore, avec les précédents votes du Sénat. Du reste, le moment venu, si la situation de l'épidémie venait à l'imposer, rien dans les textes n'empêcherait le Gouvernement de revenir devant nous après, ou même avant, le 28 février.

Cette dérogation injustifiée au secret médical nous avait déjà été proposée, dans la précipitation, en juillet dernier, et nous l'avions alors repoussée. Pour les mêmes raisons, nous estimons qu'il n'est pas judicieux de mettre en oeuvre une pareille mesure. Reconduire le dispositif actuel d'information des des responsables des établissements d'enseignement scolaire, plus global, nous paraît donc préférable. Enfin, le texte de la commission comprend un certain nombre d'autres améliorations appréciables, adoptées afin de veiller à la stricte nécessité de diverses prorogations, mais également de limiter le recours aux ordonnances. Ainsi, nos rapporteurs ont préféré supprimer du projet de loi plusieurs habilitations à légiférer par ordonnances et leur substituer occasionnellement des dispositions inscrites « en clair » dans la loi. Là encore, le Sénat est en cohérence avec sa position

Au-delà des mesures qui seront votées, et parce que nous devrons vivre encore de longs mois avec ce virus, il convient de ne pas oublier que nous disposons d'outils simples et efficaces pour nous protéger et protéger notre entourage, comme les gestes barrières ou le télétravail par exemple. Pour conclure, je salue une fois de plus l'approche pragmatique de nos rapporteurs. Partis d'un texte attentatoire aux libertés individuelles et au pouvoir législatif et de contrôle du Parlement,

Nos craintes étaient justifiées, nous le voyons bien aujourd'hui. Ce passe dessine un projet de société, un modèle social que nous redoutons et que nous dénonçons. Sous prétexte, donc, que le passe sanitaire protège et protégera, vous nous demandez de reconduire cette boîte à outils dont l'efficacité en tant que telle, c'est-à-dire le simple pouvoir de limiter l'accès des personnes non vaccinées ou non testées à certains lieux de vie, est peu étudiée et encore moins évaluée à moyen terme.

Ce que nous savons d'ores et déjà, c'est que les personnes les plus fragiles, le public prioritaire, ne sont toujours pas totalement vaccinées et que les plus précaires, les plus éloignés de l'épicentre de notre vie sociale, ne le sont pas suffisamment, âgées de plus de 80 ans ont un schéma vaccinal complet, et que le passe sanitaire n'aura sûrement aucun effet protecteur sur ces populations. Parlons des doses maintenant.

Depuis le début de la crise, l'état d'urgence a été renouvelé à plus de dix reprises. Ce projet de loi franchit une nouvelle étape : il crée un état d'urgence de précaution face à un risque non évalué.

Quant à la territorialisation introduite comme une sorte de compromis par la commission des lois, elle ne nous paraît pas non plus adaptée. Les bassins de vie et, donc, les possibles contaminations n'ont souvent rien à voir avec les frontières administratives, qu'il s'agisse des

du virus. Nous, sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, en appelons à des mesures fortes dès maintenant pour aller vers les populations non vaccinées, à des annonces claires d'une troisième dose, et ce sans lien avec une possible désactivation du passe sanitaire actuel, à un rappel énergique de l'importance des mesures barrières. Tout cela ne nécessite ni prolongation de l'état d'urgence ni maintien du passe sanitaire. C'est pourquoi nous voterons contre ce texte, contre les pouvoirs concentrés entre les mains de l'exécutif, y compris après les élections du printemps 2022, contre un passe sanitaire qui assure à ce stade une moindre protection individuelle et contre une territorialisation des

des pouvoirs de police administrative exorbitants du droit commun. Ces divers régimes juridiques, soit d'état d'urgence, soit d'état d'urgence en demi-teinte, ont conduit à une limitation des libertés individuelles et collectives sans précédent liberté de mouvement, liberté de manifester et même, à un moment donné, droit à un procès équitable. Aujourd'hui, le Gouvernement nous propose, pour l'essentiel, de proroger l'application du régime de gestion de la crise sanitaire et du passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, et de reporter la date de caducité du régime de l'état d'urgence sanitaire à la même date.

Selon nous, si le texte de la commission est bien plus mesuré que celui du Gouvernement- preuve en est la suppression des dispositions visant à créer un traitement spécifique des données de santé dans les établissements scolaires -et s'il est nettement plus respectueux de la représentation nationale, puisqu'il prévoit un contrôle de l'action de l'exécutif digne de ce nom, il n'en demeure pas moins qu'en prolongeant la possibilité de recourir à de tels dispositifs le Gouvernement, comme la majorité sénatoriale, continue à privilégier une approche sécuritaire de la gestion de crise et fait le choix de proposer une politique disciplinaire désormais banalisée au nom de la prévention sanitaire.

le rapporteur, je vous remercie tout d'abord d'avoir rappelé le succès de la campagne de vaccination organisée par le Gouvernement avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les élus locaux. Celle-ci a permis à la France d'atteindre l'un des meilleurs taux de couverture vaccinale d'Europe. L'anticipation, la réactivité dans les commandes et la distribution des doses, la finesse du maillage territorial obtenue grâce aux sites de vaccination, le soutien financier, matériel et humain

l'évolution de la vaccination et la mobilisation du système hospitalier. Madame Di Folco, l'accès des directeurs d'établissement scolaire aux données virologiques et vaccinales est nécessaire pour fiabiliser et améliorer la campagne de dépistage et de vaccination auprès des jeunes. Nous aurons sans doute de nombreux débats à ce sujet au cours de cette séance. C'est la condition pour faire progresser et pour affiner le protocole sanitaire en place dans les écoles depuis quelques semaines, lequel vise à limiter, vous le savez, les fermetures de classes dans l'hypothèse où un ou plusieurs cas positifs

Aujourd'hui, plus de 80 % des Français âgés de plus de 12 ans sont vaccinés ; les masques et les tests de dépistage sont disponibles en grande quantité et les taux d'incidence et de positivité aux tests restent très faibles. Pourtant, le Gouvernement nous demande, au cas où, de lui donner les moyens d'imposer un reconfinement ou un couvre-feu quand bon lui semble, sans avoir à nous consulter. Shooté depuis des mois à la prise de décision non concertée et non contrôlée, voilà que le Gouvernement vient nous réclamer une nouvelle dose Mes compatriotes établis hors de France, qui vivent dans des pays où le Parlement exerce un contrôle très strict de l'action du pouvoir exécutif, me disent souvent à quel point ils sont choqués de voir que, chez nous, le Gouvernement piétine les droits du Parlement et, donc, méprise les Françaises et les Français que nous représentons.

C'est pourquoi je vous demande de faire preuve de respect vis-à-vis de nos compatriotes, en revenant sur votre intention de passer par-dessus le Parlement jusqu'au 31 juillet. La parole est à Mme Esther Benbassa,

de taux d'incidence beaucoup moins élevés qu'au plus fort de la crise. La vaccination a atteint un record : 85 % des Français, dont plus de 90 aux tranches d'âge les plus à risque, ont été vaccinés. De ce fait, il est plus raisonnable, comme l'a soutenu la commission, de restreindre le passe sanitaire aux seuls départements dans lesquels moins de 75 % de la population est complètement vaccinée. Le maintien de ce dispositif sur l'ensemble du territoire, sans véritable justification sanitaire, est attentatoire aux libertés. Comme un refrain, vous ne cessez de répéter que le passe sanitaire obligatoire pousse à la vaccination massive et que l'objectif sera très bientôt

des interdictions décidées par décret. Vous semblez nier les problèmes à venir pour les élections présidentielle et législatives : y aura-t-il besoin d'un passe pour aller voter ? À quelques mois de ces échéances, vous devriez faire preuve de davantage de clairvoyance dans vos décisions. En juillet dernier, la Défenseure des droits a appelé de ses voeux l'organisation d'un débat démocratique public. Je soutiens cette initiative qui permettrait d'éclairer les zones d'ombre entourant la prorogation de ce passe sanitaire. Je reçois, comme mes collègues, des centaines de courriels de familles en souffrance, qui sont réellement touchées

Quels que soient les efforts consentis par la commission des lois du Sénat pour prendre en compte les inquiétudes légitimes de nombre de nos concitoyens, d'observateurs et d'acteurs de la vie publique et politique, nous n'approuvons pas cette version du texte.

n° 67. Nous réitérons notre opposition à la prorogation du régime juridique d'exception, qui renforce considérablement les pouvoirs de l'exécutif et qui vient normaliser et banaliser des mesures exorbitantes du droit commun. Le contrôle et la limitation stricte dans le temps de l'état d'urgence sanitaire sont essentiels,

présenter l'amendement n° 83. Je voudrais reprendre à mon compte la formule de la plus éminente de nos collègues de l'Assemblée nationale, car elle résume assez bien la situation : « Soit le vaccin est efficace et le passe ne se justifie plus

maintenant. Nous avons trop reculé ! Dans ce texte, la droite sénatoriale propose de ne proroger le passe sanitaire que jusqu'au 28 février. Quels grands seigneurs ! ! À force de compromis permanents, son refus de l'opposition vire à la compromission, à un soutien qui ne dit pas son nom. La droite sénatoriale refuse le combat avant de l'avoir commencé ! L'exécutif trinque à votre santé, à la santé de l'opposition docile

une grande vigilance s'impose face au risque d'apparition d'un nouveau variant, que nous ne pouvons prévoir aujourd'hui, et dont les caractéristiques pourraient être différentes de celles que nous connaissons déjà. Dans ce contexte qui demeure donc incertain, il est indispensable de prolonger, jusqu'à l'été, les outils de gestion

d'urgence sanitaire, défini par la loi du 31 mai 2021, et le passe sanitaire ont démontré leur efficacité pour contenir la circulation du virus, limiter les conséquences de cette circulation sur la population et sur le système de santé, tout en permettant à la vie économique et à la vie sociale de notre pays, de nos concitoyens, de se poursuivre. Si je suis favorable à un encadrement plus strict du passe sanitaire, j'estime, comme les députés, que cet encadrement doit reposer sur la prise en compte de plusieurs critères- et non pas d'un seul

Gay, je vous demande des excuses. Nos maires, et pas seulement les maires communistes- je pourrais citer d'autres formations politiques -, ont utilisé tous les outils à leur disposition pour que nos concitoyennes et nos concitoyens soient vaccinés.

un passe sanitaire pour accéder aux établissements accueillant des personnes vulnérables dans l'ensemble des départements. Les personnes accueillies dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ont fait partie des publics prioritaires pour l'accès à la vaccination. Elles sont donc majoritairement vaccinées. Néanmoins, leur extrême vulnérabilité exige de prendre un maximum de précautions : il faut à tout prix leur éviter une exposition au virus. Une contamination, même minime, peut avoir des effets redoutables, compte tenu des multiples facteurs de comorbidité

Alors que les équipements de protection individuelle sont aujourd'hui largement répandus, que nous disposons de l'une des meilleures couvertures vaccinales d'Europe et que la circulation du virus est globalement contenue, on persiste à vouloir nous accoutumer à un état d'urgence permanent qui, peu à peu, prend la place de la démocratie pleine et entière.

de remplacer le taux de 75 % par 70 %. Pourquoi 70 % ? Il s'agit, certes, d'un amendement de repli, mais ce chiffre correspond en réalité à 90 % de la population de plus de 18 ans.

Aujourd'hui, le virus SARS-CoV-2 tend à devenir endémique. Or un taux d'incidence non défini ne renseigne pas finement sur la nature de la circulation virale, non plus que sur l'apparition de la maladie. D'une part, le taux de positivité des tests de dépistage renseigne sur la présence d'un génome de virus et non d'un virus viable et infectieux. Un test de dépistage dissocié d'une symptomatologie de maladie ne donne pas d'indication sur la situation épidémiologique. Le système dit « Sentinelles » existe, mais il a été mis de côté dans le pilotage de la situation sanitaire depuis des mois, ce qui est inadmissible. De plus, le taux de positivité présente deux limites le nombre de tests réalisés et le dénominateur commun. Dans le cadre d'une épidémie, seul le rapport du nombre de cas positifs sur le nombre d'habitants peut être représentatif. D'autre part, la couverture vaccinale est indépendante de la positivité aux tests de dépistage et de la pathologie.

indépendamment de la couverture vaccinale. La vaccination avec les produits actuellement proposés n'est pas un indicateur de la situation épidémique ou de sa maîtrise. Le passe sanitaire ne se justifie donc

Les exemples de ce type sont très nombreux, générant des frustrations et un sentiment profond d'injustice. Au-delà de ces incohérences, cet amendement vise à interdire le passe sanitaire pour les mineurs pour des questions de santé et d'éthique, conformément aux préconisations du Comité consultatif national d'éthique. Son président, M. Jean-François Delfraissy déclarait ainsi le passe sanitaire ne devait pas concerner les adolescents et les enfants : « Le recul existant ne permet pas d'assurer la pleine sécurité de ces nouveaux vaccins chez l'adolescent. [ ...] Les conséquences de la pandémie sur la santé psychologique et mentale des enfants, et surtout des adolescents, sont profondes et probablement durables. S'agissant de l'immunité collective, est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes de bénéfice collectif, du refus de la vaccination d'une partie de la population adulte ? » Pour toutes ces raisons, il convient de mettre un terme au passe sanitaire pour les mineurs.

Contrairement aux secondes, toutefois, les mineurs, qui sont des citoyens en devenir ayant besoin d'interagir pour se construire, sont les moins vulnérables à l'épidémie. En effet, dans cette tranche d'âge, le taux de cas graves suivis médicalement est inférieur à 1 % et le taux de décès frôle 0 %. Dans le même temps, la couverture vaccinale à 85 % de la population est suffisante pour protéger les adultes. Il est temps de rendre à chacun la maîtrise de sa santé, en collaboration avec son médecin et son pharmacien. Continuer dans l'incitation à la vaccination des enfants, par l'obligation du passe sanitaire pour les 12-18 ans, décrédibiliserait fortement la parole politique. Pour ces raisons, cet amendement vise à sortir les mineurs des dispositifs liés au passe sanitaire.

culturelles. D'une part, le taux de vaccination des 12-18 ans est déjà très élevé, et, d'autre part, le vaccin n'a pas démontré d'efficacité totale dans la lutte contre la transmission du virus. Aussi, il n'est plus nécessaire aujourd'hui de prolonger la pression vaccinale. Par ailleurs, plusieurs études récentes font état de risques avérés de complications cardiaques chez les jeunes de moins de 18 ans. Le Parlement n'a reçu aucune information de la part du Gouvernement sur l'intégration de la troisième dose au passe sanitaire. Qu'en sera-t-il ?

Ainsi, des adolescents en surpoids pourraient, par exemple, être contraints de recevoir une troisième injection pour conserver leur passe. Or il est inacceptable d'envisager une telle mesure, non seulement discriminante, mais aussi dangereuse pour la santé mentale et physique des adolescents. Cette catégorie atteint déjà un taux de vaccination élevé, tandis que la stratégie sanitaire du Gouvernement a échoué depuis huit mois à aller vers 2,2 millions de personnes fragiles.

et à le réserver à celles qui se tiennent en lieu clos. Les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estiment que, en période de maîtrise de l'épidémie, les activités de plein air doivent rester accessibles à tous et dans les mêmes conditions. Il s'agit notamment de recréer du lien social, là où il a été brisé, tout en continuant à assurer une lutte efficace et raisonnée

C'est précisément l'objet de cet amendement. Par ailleurs, ses auteurs tiennent à rappeler qu'une telle limitation de l'application du passe sanitaire ne doit empêcher ni le respect des gestes barrières ni le port du masque, qui reste obligatoire.

au sein d'une association sportive ou d'un club, sans avoir à présenter de passe sanitaire. La pratique sportive est un élément majeur pour la santé publique de nos concitoyens. La crise sanitaire a profondément affecté la pratique des Français, notamment des plus jeunes. Le renforcement de la sédentarité est un véritable problème de santé publique, qu'il convient de combattre vivement. Par ailleurs, les retours concernant les inscriptions dans les associations sportives en ce début d'année montrent que les mineurs de 12 à 18 ans se sont éloignés de la pratique, quand le retour en club des moins de 12 ans est extrêmement dynamique.

Le service public des bibliothèques est reconnu comme essentiel, et la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, récemment adoptée par l'Assemblée nationale et en cours de navette parlementaire, reconnaît l'importance de ces lieux. Des villes ont d'ores et déjà fait le choix d'exempter l'accès aux bibliothèques de contrôle du passe sanitaire, si cela se fait dans le cadre scolaire ou universitaire. Afin d'offrir un accès libre à la culture à tous les jeunes, il convient d'exempter les mineurs de tout contrôle sanitaire pour l'accès à ces espaces de culture. L'amendement n° 60, présenté

des enfants et des adolescents. Au vu de la situation sanitaire actuelle, et dans le cas où les gestes barrières sont respectés dans ces établissements, il ne nous semble nullement nécessaire de conditionner leur accès à la présentation d'un passe sanitaire pour les mineurs de plus de 12 ans.

Il s'agit d'écarter les terrasses de cette obligation, et cela pour deux raisons simples. Premièrement, le taux de vaccination complète de la population s'est largement accru depuis quelques mois, et nous nous en félicitons. La France a été propulsée à la deuxième place au niveau européen pour le nombre de doses administrées et à la neuvième place pour le pourcentage de population complètement vaccinée. Deuxièmement, l'exigence de présentation d'un passe sanitaire représente une charge supplémentaire considérable pour les restaurateurs, qui n'ont pas toujours les moyens matériels ou humains pour en assurer le contrôle. Cet état de fait aboutit inévitablement à des situations où des établissements ne sont pas en capacité de faire respecter cette obligation, se mettant malgré eux en porte-à-faux avec les obligations légales en vigueur. Encore une fois, les taux de transmission étant nettement inférieurs en milieu ouvert, les membres de notre groupe souhaitent améliorer le texte et restreindre le recours au passe sanitaire à l'essentiel.

Le Gouvernement et l'Assemblée nationale ayant, à plusieurs reprises, balayé l'inscription de jauges applicables au passe sanitaire dans la loi, celles-ci ont finalement été fixées par décret la redéfinition de ces jauges et leur intégration dans la loi sont essentielles pour assurer la proportionnalité du dispositif que nous examinons, en particulier dans un contexte d'accalmie de l'épidémie. La jauge de 1 000 personnes

que la vaccination n'empêche pas la contamination et la transmission du virus. Aussi, cet effet pervers du passe sanitaire sur le relâchement des gestes barrières devrait nous conduire à nous interroger sur la reconduction de son usage, notamment au sein de ces milieux professionnels. Tel est l'objet de cet amendement.

aussi, que là où les gestes barrières, notamment le port du masque, sont possibles, le passe sanitaire ne soit en principe pas en vigueur, même dans les départements

L'amendement n° 5 de Mme Delmont-Koropoulis me paraît prudent. Les personnes les plus vulnérables de notre pays, même dans les départements

viens aux amendements identiques n 7 rectifié, 27 et 65, qui visent à supprimer purement et simplement le passe sanitaire. La commission a émis un avis défavorable

car c'est une condition supplémentaire posée à la prolongation du passe sanitaire dans les départements où la vaccination est en retard. Elle souhaite également que le chiffre qu'elle a retenu, qui n'est pas improvisé, soit maintenu. Ce chiffre de 75 % correspond exactement à la moyenne nationale. Vous êtes dans la moyenne nationale ou au-dessus ? Plus de passe sanitaire. Vous êtes en dessous ? Vous devrez attendre, pour que le passe sanitaire soit levé, que le taux de vaccination ait rejoint

de la population. Par conséquent, la commission a émis un avis de sagesse sur l'un de ces amendements ; elle ne souhaite pas que celui-ci soit adopté, mais elle entend se montrer conciliante.

d'incidence du virus on pourrait rétablir le passe sanitaire dans un département où la vaccination serait en retard sur la moyenne nationale. Nous nous sommes bornés à renvoyer une telle décision au Gouvernement, en mentionnant un taux de circulation du virus

il y a quelques mois, nous avons été convaincus que, même si le risque vital pour les mineurs de 12 ans à 18 ans était évidemment

un mineur contagieux peut contaminer autour de lui énormément de personnes. On fait des moyennes

obligatoire. Nous sommes d'ailleurs fermes sur nos principes quand il s'agit de ne pas divulguer les secrets médicaux de nos écoliers, de nos collégiens et de nos lycéens aux administrations des établissements d'enseignement. Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir renoncer à vos amendements ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

favorable. De même, nous sommes favorables à l'amendement n° 1 rectifié concernant les associations sportives qui organisent des activités dans le gymnase du collège. Quand ces activités sportives ont lieu dans le cadre scolaire, avec un professeur d'éducation physique et sportive,

ou feuilleter des magazines avec un masque. En revanche, on ne peut ni manger ni boire avec un masque, et ce critère de bon sens fait la distinction entre les lieux où le passe sanitaire continuera à être possible dans certains départements et les lieux où il deviendra impossible.

Quand vous êtes proches les uns des autres, vous vous exposez à un risque de contamination ; c'est vrai pour toutes les maladies virales et pour toutes les épidémies. Par conséquent, il ne me semble pas utile de fixer un nombre de personnes dans un même lieu : tout dépend de la surface

par la commission des lois

pour rappeler de manière plus générale les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne souhaite pas fixer dans la loi un seuil territorialisé de vaccination au-delà duquel le passe sanitaire ne peut plus être mis en oeuvre. Premièrement, ce type de territorialisation par référence à un seuil rigide

d'un schéma vaccinal complet, et ces jeunes se vaccinent de plus en plus, sans que cela pose de problème particulier. Sachez aussi, mesdames, messieurs les sénateurs,

toutes ses prévisions alarmistes, dont on change les critères pour les rendre encore plus alarmantes ? Je voudrais revenir sur la pression vaccinale qui pèse sur les enfants et les mineurs.

Si nous ne renonçons pas aujourd'hui à ce passe sanitaire, dans combien d'années allons-nous le faire ? Vous allez plonger la population dans l'incompréhension et la désespérance.

Je me souviens d'ailleurs que, en 1954, Pierre Mendès France avait annoncé qu'il se donnait jusqu'au 20 juillet pour conclure les accords de Genève. Le jour venu, ceux-ci ne l'étaient pas encore : on a donc arrêté les horloges jusqu'au matin

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

plusieurs amendements déposés à l'Assemblée nationale et au Sénat lors de l'examen des textes précédents alertaient déjà sur ce sujet. Quatre mois plus tard, le risque d'exclusion de la vie démocratique est plus grand que jamais, et nous n'avons reçu aucune garantie écrite de la part du Gouvernement. L'adoption de cet amendement permettrait d'en graver une dans le marbre. Quel

Les prolongations successives des diverses dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire tendent à nous faire oublier que ces mesures ne doivent qu'être exceptionnelles. La menace qui nous guette aujourd'hui n'est plus celle du virus. Nous apprenons difficilement à vivre avec celui-ci, disposons maintenant d'outils efficaces pour le contenir. Désormais, la principale menace qui plane est bien de s'habituer à ce régime d'exception et de le voir devenir permanent. C'est pour cette raison que je m'oppose au fait d'accorder de de nouveau au Gouvernement la possibilité d'ordonner la fermeture d'établissements recevant du public ou d'interdire la libre circulation des personnes et les rassemblements. L'évolution actuelle de l'épidémie ne justifie pas la prorogation d'un possible recours à des mesures aussi liberticides par l'exécutif. Nous devons maintenant concilier la lutte contre le virus et la protection de nos libertés. Pour cela, le Parlement doit prendre

l'avenir. Restons vigilants, pour nos libertés et pour notre démocratie Depuis le mois de mars 2020 et le début de la crise sanitaire, l'état d'urgence sanitaire a été renouvelé à onze reprises, sous des appellations diverses ! Nos institutions démocratiques sont éprouvées par les mesures restrictives des libertés prises pour gérer la propagation de l'épidémie. Pour lutter contre celle-ci, une politique de prévention sanitaire, de dialogue avec la société civile et d'actions destinées à lever la méfiance envers la parole publique et institutionnelle est plus efficace que la multiplication de mesures restrictives des libertés. le Gouvernement alterne entre des mesures de confinement et des mesures d'instauration et de prolongation du passe sanitaire. Il procède ainsi à une déresponsabilisation de la population. Le quotidien des Français se trouve entre les mains de quelques-uns, du bon vouloir du Président de la République et de quelques personnes qui siègent au conseil de défense. La vaccination faisant effet, la situation sanitaire ne justifie pas le prolongement des mesures restrictives. Selon Santé publique France, le nombre d'hospitalisations dues au covid est au plus bas et le taux de positivité est descendu à 1 %, après un pic à 5 % au mois d'août 2021. La vaccination et l'application des gestes barrières ont eu bien plus d'effets bénéfiques que les mesures restrictives appliquées depuis le mois Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande ainsi la suppression du régime d'exception autorisant le Gouvernement à prendre par décret les mesures de fermetures d'établissements et de restrictions des déplacements de la population.

des mesures exorbitantes du droit commun. Le contrôle et la limitation stricte dans le temps de l'état d'urgence sanitaire sont essentiels, afin de préserver un équilibre entre l'objectif sanitaire et la garantie de

nous pourrions subir les conséquences de l'apparition d'un nouveau variant encore plus contagieux que le variant delta. Il est donc indispensable de proroger jusqu'à l'été le cadre juridique de cet état d'urgence sanitaire,

je précise une fois encore qu'il s'agit bien uniquement de reporter la date à laquelle les dispositions fondant l'état d'urgence sanitaire disparaîtront de l'ordonnancement juridique. Il faudra évidemment toujours un décret en conseil des ministres pour déclarer l'état d'urgence sanitaire, et sa prorogation au-delà d'un mois,

aux personnes vaccinées d'être protégées, la question de la troisième dose devrait être examinée objectivement. Je ne vois d'ailleurs pas comment le Gouvernement pourrait l'imposer du jour au lendemain

d'imposer la présentation d'un document apportant toute garantie que la personne n'est pas contaminante, dans le cadre du franchissement des frontières. Ce dispositif a été institué jusqu'au 30 juin prochain. Les instances de l'Union européenne devront délibérer de son éventuelle prolongation. Nous devons, c'est notre engagement européen, continuer à l'appliquer jusqu'au 30 juin. Par conséquent, la date du 28 février ne peut en aucun cas être retenue pour la mise en oeuvre de ce dispositif. Quant à savoir s'il serait préférable de l'arrêter au 30 juin ou au 31 juillet, je réponds qu'il vaut mieux l'arrêter au 31 juillet, pour une raison très simple : si une décision est prise à la fin du mois de juin par les instances européennes, il faudra laisser le temps au Parlement français d'en délibérer. Or l'Assemblée nationale sera alors en plein renouvellement